Elle consacre près d’un tiers de son PIB aux prestations sociales, un niveau exceptionnel à l’échelle internationale. Ce modèle social est un pilier de notre République : il garantit un filet de sécurité à ceux qui en ont besoin. Mais, pour en assurer la pérennité, nous devons aussi veiller à son équilibre et à son équité. C’est dans cet esprit que cette proposition de loi vise à instaurer une condition de résidence de deux ans pour l’accès à certaines prestations sociales, sauf en cas d’exercice d’une activité professionnelle. Cette mesure est raisonnable et proportionnée, bien loin des neuf ans exigés au Danemark ou des cinq ans proposés par le Sénat dans le projet de loi Immigration en 2023. L’objectif est clair : garantir la viabilité de notre système de protection sociale tout en conservant son caractère solidaire. Notre modèle social, en effet, n’a de sens que s’il est soutenable dans la durée. Il s’agit ici non pas de restreindre l’accès aux aides, mais de poser un cadre juste et responsable. Soyons transparents avec les Français. Ce texte conditionne le versement de certaines prestations sociales, notamment l’allocation personnalisée d’autonomie, les aides au logement et la plupart des prestations familiales, à une durée de résidence en France de deux ans. Actuellement, ces aides sont accessibles aux étrangers en situation régulière sous réserve d’une résidence stable de neuf mois. D’autres prestations, comme le RSA et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ne sont pas concernées, car elles répondent déjà à des critères plus stricts ans de résidence pour le RSA, dix ans pour le minimum vieillesse. L’évolution proposée permet d’harmoniser notre système d’aides tout en assurant une meilleure adéquation avec la réalité des ressources publiques disponibles. L’un des débats soulevés en commission des affaires sociales porte sur les répercussions concrètes de cette mesure : combien de personnes seront concernées ? À ce stade, les données précises manquent, nous le déplorons. Toutefois, au delà des chiffres immédiats, cette réforme s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’efficacité et la pérennité de nos politiques sociales. Ce texte met en lumière nos engagements internationaux en matière sociale.

Si ces conventions permettent aux Français établis à l’étranger de bénéficier des mêmes prestations que les ressortissants des pays signataires, nous devons néanmoins nous interroger quant à leur pertinence. Sont elles réellement équilibrées, alors que la France est le seul pays proposant un modèle social aussi généreux ? Notre situation budgétaire impose d’aborder ce sujet avec lucidité. Ce n’est pas seulement une question financière : c’est une question de justice. L’équité entre les citoyens français et les étrangers bénéficiant de notre protection sociale est essentielle et nous devons veiller à ce que cet équilibre soit respecté. Ce texte ne constitue que la première pierre d’une réflexion plus large sur la maîtrise de nos dépenses sociales. Il pose un principe, mais, dans les faits, la disposition qu’il consacre restera une exception tant que nos conventions internationales ne seront pas réexaminées. cette réforme est une étape, mais elle doit s’accompagner d’un travail plus approfondi sur la rationalisation de notre modèle de protection sociale. Enfin, soyons clairs, cette mesure ne répond pas au problème de l’immigration illégale. La situation de Mayotte illustre bien l’ampleur des défis à relever, mais la question dépasse largement ce territoire : elle concerne l’ensemble du pays. Il nous faut une réponse globale, articulant politique migratoire, contrôle des frontières et gestion rigoureuse de nos finances publiques. Nous ne devons pas craindre un débat honnête sur ces sujets. Plus que jamais, la France doit reprendre le contrôle de ses frontières, de ses finances publiques et de ses choix stratégiques. Elle doit retrouver sa pleine souveraineté, et c’est là l’un des défis de notre époque. Cette proposition de loi est un premier pas dans la bonne direction. S’y affirme une volonté de responsabilité et de justice sociale. C’est dans cet esprit que notre groupe votera en faveur de ce texte.

tout d’abord, je tiens à remercier notre collègue Valérie Boyer, qui nous permet, avec ce texte, de reprendre le fil de débats que nous avons eus dans le passé sur la durée de résidence nécessaire en France pour obtenir le versement de prestations sociales et familiales, ainsi que du minimum vieillesse. Ces prestations étant versées aux étrangers qui n’exercent pas d’activité professionnelle, il semble légitime de demander à leurs bénéficiaires d’être suffisamment présents sur notre sol pour être associés à la vie collective et aux principes de solidarité qui la sous tendent.

de surcroît que notre Constitution permet de conditionner le bénéfice de certaines prestations sociales à une durée de résidence stable et régulière ou d’activité professionnelle. Cette proposition de loi s’inscrit donc pleinement dans notre droit fondamental.

reste l’un des pays les moins exigeants en la matière. Nos voisins tels que l’Italie, Chypre, l’Irlande, le Danemark ou encore la Grèce conditionnent le versement de leurs prestations à une durée de résidence qui peut aller, dans certains cas, Pour la parfaite information de nos concitoyens, il est utile de rappeler la liste de ces prestations qui sont acquises aujourd’hui avec neuf mois de résidence en France : la prestation d’accueil du jeune enfant ; les allocations familiales ; le complément familial ; l’allocation de logement ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; l’allocation de soutien familial ; l’allocation de rentrée scolaire ; l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; l’allocation journalière de présence parentale ; l’allocation de solidarité sujet, je veux souligner ici que le minimum vieillesse, versé sans condition de nationalité ni de travail, est de 1 034 euros par mois pour une personne seule et de 1 605 euros par mois pour un couple. Au moment où nous apprenons que le conclave sur la réforme des retraites ne mènera nulle part, les Français étant appelés à travailler bien au delà de 64 ans, je rappelle que les catégories les plus pénalisées par cette réforme, c’est à dire les femmes et les seniors mis au chômage dès 55 ans, n’auront guère plus en moyenne, alors qu’ils auront travaillé et cotisé pendant des décennies. Par conséquent, demander deux ans de résidence en France en contrepartie de ces prestations ne me paraît pas obéir à une quelconque idéologie

à l’image des femmes, dont les carrières hachées les obligent à occuper des emplois précaires au delà de 64 ans ; à l’image également des seniors, condamnés dès 55 ans au chômage, puis au RSA, alors qu’ils ne demandent qu’à travailler. De même, il faudrait être aveugle pour ne pas voir la bombe sociale du logement, qui est en train d’exploser et qui, là encore,

plus sa classe moyenne. En conclusion, j’assume sans difficulté le mauvais rôle qui est assigné à ceux qui défendent cette proposition de loi. La générosité des idéaux promus par certains est malheureusement incompatible avec la réalité vécue par la majorité des autres.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre rapporteure l’a très justement rappelé en commission la semaine dernière, la question qui se pose aujourd’hui est avant tout celle de la définition de notre modèle de protection sociale. « La sécurité sociale n’est pas une charge, c’est un investissement dans la dignité humaine », disait Pierre Laroque, l’un de ses fondateurs. C’est une promesse : celle d’une République solidaire qui protège chacun de ses résidents face aux aléas de la vie.

Ce texte reprend l’esprit d’un amendement introduit au Sénat dans la loi Immigration. À l’époque, Marine Le Pen s’était félicitée de cette mesure : elle y voyait une « victoire idéologique du Rassemblement national » et la consécration de l’idée de « priorité nationale » que son parti défend depuis plus de quarante ans. Absolument ! Est ce vraiment cette direction que nous voulons suivre ? On nous explique qu’il s’agit de limiter l’appel d’air migratoire produit par un régime social qui attirerait l’immigration illégale. Mais où sont les chiffres qui le prouvent ? Aucune étude ne démontre qu’une telle mesure aurait un quelconque effet sur les flux migratoires. Prétendre que la France est un eldorado social dont les aides attireraient les étrangers, c’est relayer une fausse idée. Les migrations sont avant tout motivées par l’emploi, et non par les prestations sociales. De la même façon, nous savons que cette proposition de loi n’aura aucun effet budgétaire significatif. La logique économique de ce texte est même contestable. Les prestations sociales doivent être vues non pas comme une charge pesant sur l’économie, mais plutôt comme un outil d’investissement social permettant la réduction des inégalités et favorisant la participation à la vie économique. un système de protection sociale qui fonctionne renforce la cohésion sociale et améliore la situation économique d’un pays, en lui évitant les coûts liés à la grande pauvreté et à la marginalisation.

en revanche, c’est que ce texte risque d’accroître la précarité de personnes qui sont en situation régulière sur notre territoire, et ce au mépris de nos principes républicains. Refuser ces aides à des personnes qui en ont besoin, c’est les précipiter dans la pauvreté, les empêcher de s’insérer durablement dans notre société. Refuser ces aides revient également à accroître le recours aux aides d’urgence, ce qui pèsera,, sur d’autres dispositifs publics et sur les collectivités territoriales. Au delà des arguments que je viens d’évoquer se pose la question de la portée de cette proposition de loi, qui semble plus que limitée. Elle repose sur une illusion d’efficacité. Différents organismes de protection sociale, mais aussi la direction de la sécurité sociale, ont relevé

Dans ces conditions, j’avoue ne pas comprendre cet acharnement de nos collègues à vouloir faire adopter un dispositif inapplicable… Mes chers collègues, l’intégration ne se décrète pas, elle se construit. Mais comment peut on s’intégrer dans un pays qui commence par vous dire « attendez deux ans avant d’être traité comme les autres » Certes, nous devons être responsables dans notre approche des politiques sociales et migratoires. Mais la responsabilité, ce n’est pas stigmatiser une partie de la population, ce n’est pas priver certaines familles d’aides essentielles, ce n’est pas affaiblir le principe d’égalité devant la solidarité nationale. J’y insiste, notre système de protection sociale est un pilier de notre pacte républicain. Il ne doit pas être instrumentalisé pour flatter des peurs et nourrir des divisions. Parce que ce texte est profondément contraire à nos principes de justice sociale et de cohésion nationale, le groupe du RDSE votera contre dans sa très grande majorité. La parole

Madame la présidente, madame la ministre,

Cette proposition, présentée par notre collègue Valérie Boyer, que je salue, vise à établir une durée minimale de résidence de deux ans pour les étrangers en situation régulière souhaitant bénéficier de plusieurs aides sociales, sauf s’ils exercent une activité professionnelle. Cette question de la conditionnalité de nos prestations sociales, ou plutôt l’idée d’exiger un temps de présence minimale sur le sol français

C’est une manière de tourner définitivement le dos à une immigration trop longtemps subie. Si cette remise en cause est largement souhaitée par l’opinion française, elle ne va naturellement pas de soi pour tout le monde. Ainsi, certains peuvent douter de l’efficacité des mesures proposées et de la réalité des effets de cette

La réalité démographique est implacable. Les taux de natalité extrêmement élevés en Afrique subsaharienne, conjugués à l’extrême pauvreté bien triste de ces pays, peuvent entraîner des mouvements de population massifs vers l’Europe et vers la France. Il est donc responsable et indispensable d’envoyer un signal aux populations de ces pays

avancés par les auteurs du texte repose sur la nécessité d’assurer un accès équitable aux aides sociales. Aujourd’hui, plusieurs de ces prestations, comme les allocations familiales ou les aides au logement, ne requièrent qu’un titre de séjour en cours de validité et une résidence de quelques mois. Cette situation est parfois perçue comme une incitation à l’installation immédiate sur notre territoire, sans véritable lien avec l’effort contributif. En introduisant une durée de résidence minimale, nous affirmons un principe l’accès aux prestations sociales doit être lié à une certaine stabilité sur le territoire national. Il s’agit d’une mesure qui existe déjà dans d’autres pays européens. Le Danemark, par exemple, exige six ans de résidence

encadre strictement les prestations sociales versées. Il n’est pas illogique, au moment où il va falloir demander des efforts pour réguler nos dépenses sociales et diminuer nos déficits, que nous cherchions aussi à réguler l’accès à nos prestations sociales. Même si le périmètre exact

Je le redis, cette mesure est conforme aux principes constitutionnels. Certains opposants à cette réforme avancent qu’elle pourrait être discriminatoire ou contraire aux principes fondamentaux du droit.

constitutionnels. Il a néanmoins jugé que la proposition initiale de fixer cette durée à cinq ans était disproportionnée. En l’abaissant à deux ans, et en excluant les travailleurs, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire,

la sécurité juridique du texte. Ainsi, nous avons remplacé la condition de « résidence stable » par l’exigence d’être titulaire depuis deux ans d’un titre de séjour, ce qui permet une vérification plus fiable des critères d’éligibilité. Nous avons également exclu le droit au logement opposable du champ d’application du texte afin de ne pas remettre en cause un principe à valeur constitutionnelle. En réalité, ce texte est aligné avec nombre de pratiques européennes. La France ne fait que se conformer à ce qui existe ailleurs en Europe. La plupart de nos voisins conditionnent l’accès aux prestations sociales à une certaine durée de résidence ou d’activité : cela n’a rien de scandaleux. Loin d’être une mesure isolée, cette réforme s’inscrit donc dans une tendance générale visant à concilier accueil et intégration responsable. Bravo ! Comme je l’ai souligné précédemment, Enfin, ce texte vise à répondre à une préoccupation croissante de nos concitoyens : celle de maîtriser les flux migratoires et de lutter contre l’effet d’attractivité que peut exercer notre système social. Pour conclure, mes chers collègues,

je vous remercie,

à deux ans. En commission des affaires sociales, nous vous avons interrogés pour connaître le nombre de potentiels bénéficiaires après cet allongement du délai de résidence : vous n’avez pas pu nous répondre.

les engagements internationaux de la France et contrevient aux principes mêmes de notre modèle social. Là aussi, ce n’est pas ce qui vous importe. Ce qui importe à la majorité sénatoriale, c’est d’occuper le terrain de l’immigration en tenant un discours radical à la place du Rassemblement national, quitte à perdre des électeurs humanistes, rationalistes et gaullistes sociaux.

Derrière l’instauration d’un délai de carence de deux années pour accéder aux prestations sociales, vous aggravez la précarité, le nombre de travailleurs pauvres et de mal logés. Selon l’Union sociale pour l’habitat (USH), cette mesure jette des ménages dans les bras des marchands de sommeil,

contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), ces délais de résidence vont restreindre les droits et engendrer une hausse de la précarité. Cette proposition de loi sonne donc comme une victoire idéologique pour le Rassemblement national auquel vous reprenez le mythe de l’appel d’air et le principe de préférence nationale. Jordan Bardella ne s’exprimait pas autrement lorsqu’il disait que « notre pays doit cesser d’être un guichet social pour l’immigration du monde entier ». Après avoir imposé l’austérité budgétaire sur les peuples, la mise en concurrence des travailleurs, voilà la phase suprême du capitalisme, qui consiste à justifier l’instauration d’une sécurité sociale à deux vitesses. remettre en cause l’universalité des prestations sociales, déjà affaiblie depuis 2016 avec le conditionnement des prestations familiales à six mois de résidence Finalement, entre ceux qui ont voulu réduire les dépenses sociales en limitant les droits des étrangers et ceux qui ont voulu réduire le nombre d’étrangers pour diminuer les dépenses sociales, il y a un point commun, à savoir la remise en cause de notre modèle social auquel, pour notre part, nous sommes profondément attachés. En généralisant et en allongeant les délais à deux ans, vous remettez en cause le principe même de l’universalité des prestations non contributives. Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons bien évidemment contre ce texte.

Monge. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la proposition dont nous débattons est une troisième tentative d’inscrire dans la loi une mesure déjà censurée deux fois par le Conseil constitutionnel. Le législateur prend sciemment un risque constitutionnel. S’il insiste, c’est d’abord et surtout pour faire entrer dans le débat, à force de répétition et à défaut de vérité empirique et scientifique, le concept d’appel d’air

du principe de proportionnalité, qui n’est pas réductible à un quantum, mais qui doit répondre aussi du caractère nécessaire et adapté d’une mesure portant atteinte à des droits fondamentaux. De surcroît, l’introduction d’une exception d’opposabilité au titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler dans le seul but de sécuriser cette proposition de loi en consentant aux exigences du droit européen reste sans aucun rapport avec l’objet des prestations concernées. Il faut toujours respecter le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe posé selon lequel « tout être humain […] a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Lorsqu’il était président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, qui a siégé dans cet hémicycle, avait déposé sur son bureau l’affichette suivante : « Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise. Mais toute loi mauvaise n’est pas nécessairement anticonstitutionnelle. » Vous faites fort, parce que cette proposition de loi nous semble répondre aux deux critiques : potentiellement inconstitutionnelle et assurément mauvaise ! Elle prend ancrage dans une récurrence de restrictions des droits des personnes étrangères, même en situation régulière, pour satisfaire un parti ouvertement Cette proposition de loi est d’abord un outil de communication politique. Faute de pouvoir imposer la condition de nationalité dans l’ensemble du champ de la protection sociale et au fur et à mesure que l’immigration a été désignée en France comme un problème public, les droits ont été soumis à une condition de résidence, puis à une condition de résidence régulière et enfin à une condition d’antériorité de séjour régulier, qui s’apparente à une préférence nationale déguisée. Ce mouvement s’accompagne de la multiplication d’obstacles administratifs, se traduisant par des renvois fréquents à des situations irrégulières après une période en situation régulière et donc à des ruptures de droits. Il s’agit d’exclure le plus de personnes étrangères possible de l’accès aux prestations sociales. Le texte alimente une triple rupture d’égalité. La première, qui existe entre les nationaux et les étrangers, s’élargit. La deuxième s’introduit entre les étrangers présents depuis au moins deux ans et les autres. La troisième s’applique au regard des prestations sociales visées ou non par la proposition

les droits des étrangers en situation régulière sont attaqués. C’est bien la figure de l’étranger qui est visée. Or être hostile par principe aux étrangers, même en situation régulière en France, doit être qualifié, car refuser de nommer

En ciblant les étrangers, c’est l’ensemble de la société qui s’abîme. D’abord, parce que cette proposition de loi entraînera une dégradation des conditions d’existence et une paupérisation des étrangers régularisés depuis moins de deux ans ou qui ne seront pas en mesure de prouver les deux ans de résidence régulière.

Dans un avis de janvier 2024, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pointait « l’inéluctabilité l’inéluctabilité de l’augmentation et de l’aggravation de la pauvreté des étrangers du fait des restrictions des conditions d’éligibilité aux prestations sociales

et de cet article, tiré de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Introduit en séance par voie d’amendement, ce dispositif a été censuré une première fois par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’il n’avait pas de lien avec le texte initial. Il a été une seconde fois censuré dans le cadre du projet de référendum d’initiative partagée, déposé par le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, les sages considérant cette fois que la durée de présence minimale envisagée était « disproportionnée Plusieurs propositions de loi se sont succédé depuis, dont le texte que nous examinons aujourd’hui. Sans suspense, mon groupe est en désaccord sur le fond comme sur la forme. Ce texte tend à instaurer une durée minimale de résidence pour les étrangers extracommunautaires en situation régulière de deux années avant l’accès aux prestations sociales, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à l’aide personnalisée au logement. Le texte prévoyait initialement de restreindre le droit au logement opposable : cette mesure a été justement supprimée en commission, le droit à un logement décent étant reconnu comme objectif à valeur constitutionnelle. Le conditionnement des prestations à une durée de séjour existe déjà. Vous avez cité le revenu de solidarité active, dont le bénéfice exige une présence sur notre sol de cinq ans. C’est également le cas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans les faits, il existe bel et bien une obligation de durée de résidence de neuf mois pour bénéficier des prestations familiales. Instaurer une carence de deux ans pour les étrangers extracommunautaires en situation régulière ne travaillant pas est il réaliste dans ce contexte ? bilatérales de sécurité sociale que la France a signées avec de nombreux pays, il est permis d’en douter. Au motif de décourager la venue des personnes étrangères au nom de la théorie de l’appel d’air, que réfutent tous les travaux sur le sujet, les mesures de ce texte tendent à remettre en cause le principe d’universalité. N’ayons pas peur de le dire : ce texte cultive l’idée d’une France méfiante, refermée sur elle même, incapable de tendre la main.

qui résident dans notre pays, qui sont en situation régulière et qui cotisent pour notre système social commun. En réalité, la suppression de ces aides sociales pour certains ménages aura une conséquence directe : l’aggravation de la pauvreté et la détérioration des conditions de vie de ménages déjà précaires. Au delà d’une constitutionnalité incertaine, ce texte risque surtout d’être inapplicable, car contraire aux conventions bilatérales que notre pays a signées. Celles ci contiennent des clauses dites de réciprocité. Cela signifie concrètement que la France s’engage à traiter les ressortissants des pays parties aux traités de la même manière que ses ressortissants concernant l’accès à la sécurité sociale.

étrangers en situation régulière originaires de ces pays ne seraient donc pas concernés par ces dispositions. Quant à la « cohérence politique » avancée pour justifier le vote de cette proposition de loi, elle ne nous apparaît pas aussi clairement qu’à vous, mes chers collègues. J’ajoute

Gouvernement a érigé la lutte contre l’immigration irrégulière au rang des priorités de notre action diplomatique. Nous soutenons cette voie et nous nous réjouissons que la délivrance des visas puisse enfin tenir compte de la qualité de la coopération migratoire des pays d’origine, s’agissant en particulier

la contribution concrète des étrangers à l’économie de notre pays.

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, vous nous avez habitués à divaguer régulièrement sur les étrangers en situation irrégulière. Cette fois, vous vous attaquez aux étrangers en situation régulière. Je ne m’attarderai pas sur les arguments juridiques, d’autres le feront mieux que moi. C’est l’aspect moral de ce texte qui me choque. La France est historiquement le pays des droits de l’homme, un phare social et universaliste. Or, depuis plusieurs mois, vous œuvrez à rendre le pays hostile à l’autre. On se demande à chaque fois quelle sera la prochaine étape, quel sera le prochain recul social : force est de constater que votre ingéniosité ne nous déçoit jamais Dans ce que vous appelez une logique de prévention de l’immigration irrégulière, vous repoussez encore un peu plus les limites de l’acceptable. Je veux bien admettre toute l’utilité de la prévention dans de multiples politiques publiques, mais pas sur ce sujet. Cela ne peut se faire en privant de droits sociaux une partie de la population.

la part des ménages étrangers ne percevant aucune ressource est passée de 42 % en 2013 à 52 % en 2023, soit une hausse de dix points en dix ans. Les ménages étrangers en situation régulière sont deux fois plus nombreux – soit 40 % – à ne pas recourir

94 % des ménages français. Enfin, 84,6 % des personnes de nationalité étrangère vivent dans un logement précaire. L’article 1 privera des familles entières du bénéfice des allocations familiales, du complément familial, des allocations de soutien familial, des prestations d’accueil du jeune enfant, des allocations d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation journalière de présence parentale et de l’allocation versée

sans explication logique ou cohérente. Inclusions et exclusions paraissent totalement discrétionnaires. L’APA est visée par cette proposition de réforme, mais pas la PCH. Pourquoi ?

Un ressortissant étranger, bien qu’en situation régulière, ne pourrait bénéficier des APL qu’après deux ans de résidence si ce texte était adopté et entrait en vigueur.

Il résultera de tout cela un système kafkaïen, dans lequel un étranger bénéficiant des APL au titre de son statut d’étudiant en perdra le bénéfice à l’issue de ses études s’il ne possède pas immédiatement un titre de séjour l’autorisant à travailler.

quel que soit leur statut migratoire, doit être considérée. Limiter l’accès à cette aide fragiliserait davantage les populations âgées déjà en difficulté et irait à l’encontre des principes d’inclusion et de solidarité sur lesquels repose notre modèle social. Je regrette aussi l’absence

qui peut défendre l’idée qu’une personne âgée dépendante devrait attendre deux ans avant de pouvoir être accompagnée ? Pourquoi une personne âgée ne serait elle pas aussi légitime dans sa demande d’accompagnement qu’une personne en situation de handicap,

Ne serait ce que pour cette raison, j’espère que cette inégalité devant des prestations de même nature, selon votre bon vouloir, sera censurée.

Cette proposition de loi repose sur l’idée que la générosité d’un système social exposerait le pays à un afflux d’étrangers. Selon encadrer strictement l’accès aux prestations sociales contribuerait à limiter leur venue sur le territoire et à les dissuader d’entreprendre le voyage. Mais

de tirer de telles conclusions ? D’un point de vue économique, la population immigrée a un effet positif sur les finances publiques. Pourtant, vous persistez à vouloir créer deux niveaux de droits entre les Français et les étrangers. Cette préférence nationale oppose nos concitoyens sur des bases xénophobes et rompt avec les principes de notre sécurité sociale. En 1945, à la Libération, notre pays a construit une sécurité sociale qui reposait sur l’idée que toute exclusion fondée exclusivement sur la nationalité devait disparaître. Pierre Laroque disait qu’il fallait considérer « l’homme, l’individu, la famille en eux mêmes […] en faisant de plus en plus abstraction de leur pays d’origine, pour leur assurer le bénéfice de toutes les garanties sociales prévues par la législation du pays où ils travaillent ou vivent ». L’universalité des prestations sociales est un fondement de notre ciment républicain. Accentuer les différences, comme vous le proposez,

Oui, la protection sociale est l’expression de la solidarité nationale. Oui, la mise en place d’une durée de résidence préalable au bénéfice de prestations sociales est souhaitable. C’est donc fort de ces convictions que nous voterons ce texte.

Et pourtant, voilà plusieurs semaines que nous discutons de textes qui remettent en cause notre universalité et notre humanisme. J’ai écouté le débat depuis le début. Je m’adresse avec beaucoup de respect à mes collègues de droite

de « préserver les conditions de bon fonctionnement des mécanismes des prestations sociales », vous savez très bien ce que vous faites : vous montrez du doigt, vous jugez des étrangers, vous allez juger des Français, trier les bons et les mauvais, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les Européens, les extra Européens, vous allez trier les familles et trier au sein même des familles. Quant à vous, madame la ministre, franchement, votre appel à la sagesse est un égarement, une inconscience

de l’universalité et de l’humanisme de notre modèle social.

La France n’est pas le Danemark ou la Grèce ! Ces pays ne sont ni racistes ni xénophobes. Ils font partie de notre bien commun européen et certains sont même socialistes…

Mme Lassarade, qui disait : « La protection sociale est l’expression de la solidarité nationale : conditionner son accès à une durée de présence en France, c’est au fond considérer que c’est l’appartenance au collectif et la participation à la vie de la Nation qui fondent la légitimité de cette solidarité. » Je vous